prises pour son application, la commission des affaires économiques a émis un avis favorable- 21 voix pour, 1 voix contre -à la reconduction de Mme Élisabeth Ayrault aux fonctions de présidente du directoire de la Compagnie nationale du Rhône. J'informe le Sénat que des candidatures ont été publiées pour siéger au sein des éventuelles commissions mixtes paritaires chargées d'élaborer un texte commun, d'une part, sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2017-157 du 9 février 2017 étendant et adaptant à la Polynésie française certaines dispositions du livre IV du code de commerce relatives aux contrôles et aux sanctions en matière de concurrence et, d'autre part, sur le projet de loi pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie. Par ailleurs, j'informe le Sénat que la commission des lois propose des candidatures pour siéger au sein de la commission mixte paritaire sur la proposition de loi visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier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 L'ordre du jour appelle la nomination des vingt et un membres de la mission d'information sur la pénurie de médicaments et de vaccins, créée sur l'initiative du groupe Les Indépendants-République et Territoires en application du droit de tirage prévu par l'article 6 du règlement.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 heure. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous

le point important de ce texte, le titre I et l'article 1, celui que vous avez voulu mettre en avant comme l'inversion de la construction du prix. Permettez-moi tout d'abord de vous dire, monsieur le ministre, que les États généraux

très fort ? Par exemple, l'Argentine utilise le glyphosate non réglementé ; le Brésil, le soja transgénique, le Mexique, les farines animales, ou encore l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les hormones de croissance. Alors je vous pose une question simple : est-ce que vous considérez que l'agriculture

Fait assez rare dans cette assemblée, les orientations et les objectifs annoncés font plutôt consensus : on est tous d'accord sur les objectifs. Tout le monde, même les plus libéraux, reconnaît que la main invisible du marché étrangle nos agriculteurs et qu'il est indispensable d'établir des règles pour les protéger de la concurrence. Ainsi, comme cela a été rappelé, le Gouvernement poursuit l'oeuvre des deux précédents gouvernements en étoffant une nouvelle fois le mécanisme de contractualisation mis en place par la loi de 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche, sans cesse renforcé depuis lors, sans répondre à la crise structurelle que connaît le monde agricole. Nous approuvons l'inversion du mode d'établissement des contrats, qui seront désormais proposés par le producteur et non plus par l'acheteur, ce qui constitue une véritable avancée. Dans la même logique, la prise en compte, dans les contrats, d'indicateurs relatifs au coût de production va également dans le bon sens. On regrette néanmoins, comme l'a expliqué Fabien Gay, que la loi ne précise pas la manière de les prendre en compte ni ne détermine d'indicateur unique à même de consolider les contrats. Le projet ne prévoit en fait aucune contrainte pour l'acheteur. même à espérer une légère amélioration de la répartition de la valeur, ce qui redonnera un peu d'air à nos paysans, mais rien n'est moins sûr. Outre ce manque d'ambition, nous déplorons vivement que ce projet ne s'attaque pas aux véritables problèmes que sont la concurrence exacerbée au sein de l'Union européenne et la multiplication des accords de libre-échange- Fabien Gay vient d'en parler -, qui exposent nos agriculteurs à la concurrence déloyale de denrées alimentaires venant du monde entier et qui sont produites dans des conditions sociales et environnementales souvent douteuses. Cette injustice sociale se double en plus d'une aberration écologique ! Pour protéger les bénéfices à l'export de quelques grands agriculteurs, on continue à exposer les autres à une concurrence délétère, qui entraîne une baisse incessante du prix de revient des agriculteurs et de la qualité de la production. Aussi, pour permettre aux femmes et aux hommes qui nous nourrissent au prix d'un dur labeur de vivre dignement de leurs productions, il faut changer de logique économique. C'était d'ailleurs l'orientation des amendements tendant à insérer un article

sur l'article. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous partageons tous ici la même volonté d'assurer une rémunération plus juste à nos agriculteurs. C'est cette volonté qui a porté les États généraux de l'alimentation et qui est la finalité principale de ce projet de loi. La rénovation du cadre contractuel pour le secteur agricole et alimentaire offre une sécurisation des débouchés, de la visibilité aux acteurs et permet, surtout, d'inverser les rapports de force en faveur de nos agriculteurs. Pour que ce dispositif soit effectif et aboutisse à un partage de la valeur ajoutée plus juste, tous les maillons de la chaîne alimentaire doivent prendre leur responsabilité et se coordonner. Le rôle confié actuellement à l'Observatoire de la formation Nous soutiendrons donc les modifications proposées par le Gouvernement, afin que l'OFPM ne soit qu'une aide apportée aux interprofessions dans leur élaboration d'indicateurs et non un palliatif à leur manque de coordination. de loi établit un cadre commun à toutes les filières, ce qui améliorera leurs relations contractuelles. Il ne s'agit donc pas d'établir d'exception pour telle ou telle filière. certains amendements qui nous sont aujourd'hui proposés visent à améliorer le dispositif présenté. Ils prévoient de conserver la liberté contractuelle et permettent de clarifier le rôle de chaque acteur dans la transformation de notre modèle agricole. Nous les soutiendrons donc. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la juste reconnaissance du travail des agriculteurs est au coeur de ce projet de loi et de son titre I. Dans mon département du Gers- j'aurais pu tout aussi bien citer d'autres exemples, l'Aude, notamment -, 109 éleveurs sont en ce moment même injustement victimes de la révision des zones défavorisées. Ils vont perdre d'ici à quelques mois la quasi-totalité de leurs indemnités compensatoires de handicaps naturels, les ICHN, une perte de 1 million d'euros sur un total de 6 millions d'euros pour le département. C'est un drame, et nous ne sommes pas là sur un cas d'école, si j'ose dire, puisque vous entendez- je partage avec vous cet objectif, monsieur le ministre -redonner de la valeur à la production. À cause de petites régions agricoles découpées il y a soixante ans- comme si les choses n'avaient pas bougé depuis lors !-les critères de révision de la carte aboutissent à des non-sens : là où l'on a toujours pratiqué de l'élevage, il faut arrêter là où l'ICHN forme la totalité ou l'essentiel du revenu de l'éleveur, on l'interrompt ! La répartition de la valeur résulte tout au long de la chaîne de rapports de force, et, avec ce texte, elle résulte directement des aides publiques, et vous avez, monsieur le ministre, le pouvoir de préserver cette valeur. Aussi, je vous suggère, avec les éleveurs, d'ajuster leurs droits à paiement de base à la moyenne nationale et d'étudier, par exemple, le classement de ces territoires en zone intermédiaire de type Piémont pour coller à la réalité, tout simplement. Je vous proposerai un amendement en ce sens. Une nouvelle fois, monsieur le ministre, je vous demande de faire et- pourquoi ne pas le dire ? -de sensibilité et même d'humanité dans la façon de gérer au mieux, et dans l'esprit de votre texte, la situation de ces éleveurs qui ne demandent qu'à vivre de leur travail et de leur vocation.

que méritent ces agriculteurs éleveurs gersois. La parole est à M. Daniel Chasseing,

Nous le savons tous, l'agriculture française est reconnue dans le monde entier pour sa diversité et son immense qualité, mais, il faut bien le reconnaître, elle est fragilisée par les crises successives- crises climatiques, sanitaires, économiques - ; d'où la nécessité d'intervenir pour, comme le prévoit le titre I, un meilleur équilibre des relations commerciales et une agriculture saine et durable. Avant la discussion de ce texte en séance publique, j'ai rencontré des agriculteurs et les syndicats de mon département : ils espèrent, monsieur le ministre, des retombées positives, même s'ils reconnaissent des difficultés d'application. Bien sûr, l'inversion du processus du prix payé aux agriculteurs est théoriquement positive. Mais il faut savoir ou avoir conscience qu'un agriculteur est obligé de vendre son produit dès qu'il est prêt à la consommation, tout simplement parce qu'il ne peut pas le conserver indéfiniment. Par conséquent, peu importe le prix, il doit s'en séparer.

le fait que l'agriculture est mondiale. Et il faudra bien sûr contrôler les grandes surfaces. C'est un premier pas. Vous devez, monsieur le ministre, interdire, en plus, l'importation de produits ayant subi des traitements proscrits en France et en Europe

ou, mieux peut-être, d'un gros rat ! Tout dans la nuance ! Les États généraux de l'alimentation ont été prolixes et ont suscité un certain espoir, mais le résultat est en grande partie décevant. Le contexte européen, nous le connaissons, puisque la Commission européenne envisage très ouvertement une baisse du budget de la PAC.

Le financement de la PAC doit non seulement garantir notre souveraineté alimentaire, mais aussi assurer une juste rémunération de ses acteurs, à commencer par les producteurs. Or la baisse du budget de la PAC se traduira, demain, par une nouvelle baisse du revenu des agriculteurs, nous le savons. C'est une lourde responsabilité, monsieur le ministre, alors que leurs revenus ne cessent déjà de s'effondrer, à tel point qu'ils ont atteint, pour certains, un niveau indécent. L'article 1, et les suivants, en traitant de la contractualisation, doit impérativement permettre une juste redistribution des marges entre les producteurs, les transformateurs et les distributeurs. Le fait même que l'on doive légiférer une nouvelle fois, cela a été dit, montre bien que les relations entre les professionnels sont aujourd'hui déséquilibrées. Les victimes de ce déséquilibre sont nos producteurs et nos éleveurs, alors que ce sont précisément eux qui nous nourrissent ! Je rappelle que, selon le dernier rapport de l'Observatoire de la formation des prix et des marges remis le 19 juin, le 19 juin, « les prix payés aux agriculteurs ont été à nouveau inférieurs à la réalité des coûts de production et n'ont pas couvert la rémunération du travail et du capital, et cela même en tenant compte des aides européennes ». La grande distribution continue, quant à elle, à conforter ses marges : cherchez l'erreur Ce télescopage d'informations et de rendez-vous européens dans notre actualité doit stimuler nos débats dans le cadre de ce texte, mes chers collègues. En inversant le mécanisme de construction des prix, en intégrant le coût des produits agricoles, il y a nécessité de revaloriser de manière concrète et significative le revenu de nos agriculteurs. Cependant, il faudra que l'État se donne les moyens de faire respecter ce nouveau cadre commercial. Pour conclure, je veux évoquer le secteur du sucre, moi qui représente ici le premier département sucrier, secteur dont le régime des quotas a pris fin en 2017 et pour lequel on constate une forte plongée des cours, comme ce fut le cas pour le secteur laitier en 2015. À cet égard, j'ai déposé un amendement tendant à renforcer la contractualisation au sein de cette filière, notamment en affermissant le rôle de l'interprofession, dans le strict respect du droit de la concurrence, assurant ainsi aux producteurs les mêmes garanties qu'aux autres agriculteurs. Très bien

par les mécanismes qu'il propose, l'article 1 est l'un des axes forts du projet de loi visant à rééquilibrer les relations commerciales entre les producteurs et les acheteurs.

Rendre l'initiative du contrat au producteur et construire le prix autour d'indicateurs prenant en compte, notamment, les coûts pertinents de la production agricole permettra- je l'espère, nous l'espérons tous -un meilleur partage de la valeur. À ce stade des discussions, le dispositif est plus équilibré qu'il ne l'était dans le projet de loi initial. L'Assemblée nationale a transféré l'émission des indicateurs aux interprofessions. La liberté qui était laissée aux parties de choisir leurs propres indicateurs n'était pas, à l'évidence, de nature à garantir des négociations sereines. Le groupe du RDSE proposera d'aller plus loin, avec l'intervention de l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Quelle que soit la voie qui sera retenue, il n'est plus admissible que les producteurs vendent en dessous des coûts de production. Aucun autre acteur économique n'accepterait de le faire ! Beaucoup d'agriculteurs ont assez souffert de la volatilité des prix et d'un rapport de force trop favorable aux centrales d'achat. Lors de la crise du lait, en 2015, dans les territoires ruraux, tous ici nous avons croisé le regard d'agriculteurs en situation de détresse, abandonnant leur exploitation, pour ne pas parler du pire. L'année dernière, le Premier ministre a conclu les États généraux de l'alimentation en souhaitant « non des compromis, mais des solutions durables ».

L'article 1 prévoit des mesures visant à modifier le cadre applicable aux contrats : si celles-ci vont dans le bon sens, elles ne seront néanmoins pas suffisantes pour assurer l'équilibre des relations commerciales. Je proposerai plusieurs amendements pour aller plus loin, notamment en vue de garantir que les indicateurs utilisés pour la formation des prix soient clairs, accessibles, transparents, équilibrés et prennent réellement en compte les coûts de production. Mais, nous le savons tous, ces mesures, même renforcées, ne seront pas suffisantes pour garantir une juste rémunération aux agriculteurs. Notre système ultralibéral, il faut le dire, fait que nous sommes limités à la fois par le droit international et par le droit européen, pour favoriser les prix à la production. La loi de 2008 de modernisation de l'économie, issue du rapport pour la libération de la croissance française, a conduit à la dérégulation. La libéralisation complète des marchés, souhaitée par les gouvernements de l'époque, en cogestion avec le syndicat majoritaire, nous amène aujourd'hui à la situation catastrophique que nous connaissons. Je continuerai à le rappeler dans cet hémicycle, à l'heure du CETA et des autres traités internationaux, il est plus que nécessaire que les produits alimentaires soient sortis, dans notre intérêt, des accords avec les autres pays du monde, notamment des pays du Sud, des accords de libre-échange et des logiques de dérégulation des marchés. Je souhaite aussi, avant d'entamer la discussion du titre I, préciser que je m'inscris en faux contre la présentation faite par certains, qui ne voient pas d'autre partie dans ce texte susceptible de concerner le revenu des agriculteurs. Le titre II serait alors une simple réponse aux demandes du reste de la société et ne serait constitué que de contraintes pour des agriculteurs déjà à bout de souffle. Cette lecture est trompeuse. La promotion d'une alimentation durable la relocalisation des productions, la sortie des pesticides, sont, elles aussi, autant de moyens pour nos agriculteurs de trouver des revenus. Ce n'est pas en tentant de regagner des parts de marché dans la compétition mondiale et en fonçant tête baissée dans la course au moins-disant social et environnemental que l'on retrouvera du revenu. C'est au contraire en développant la valeur ajoutée, la qualité la qualité et les circuits de proximité que l'on pourra assurer une transition de l'agriculture qui bénéficiera à la fois aux producteurs et à la société tout entière, sans oublier les générations futures. La La parole est à M. Guillaume Chevrollier, sur l'article. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'agriculture est un secteur stratégique pour notre pays et pour nos territoires ruraux. Avec 450 000 exploitations agricoles et 2 millions d'emplois directs, la France agricole permet notre souveraineté alimentaire. En outre, notre agriculture s'exporte partout dans le monde. Pourtant, elle est soumise à trop de charges, trop de normes, trop de contrôles. Bien plus, nos agriculteurs ne sont pas suffisamment payés de leur travail. travail. Ils attendent des solutions concrètes et pérennes depuis longtemps déjà- je l'entends régulièrement sur le terrain dans mon département, la Mayenne. Les États généraux de l'alimentation ont créé des espoirs de rémunérations plus justes. Cela devrait être notre préoccupation première. Pourtant, le projet de loi n'a pas été fidèle à cet objectif : à l'origine davantage alimentaire qu'agricole, le texte remodelé par le Sénat revient à l'essentiel, à savoir permettre aux agriculteurs de vivre décemment de leur travail, réduire leurs charges et leurs contraintes, promouvoir les productions locales de qualité. on relève plusieurs avancées visant notamment à rééquilibrer les rapports de force dans les relations commerciales, à mieux partager la valeur ajoutée, à supprimer les surcoûts de charges et de contraintes pour les agriculteurs qui ont été introduits lors des débats à l'Assemblée nationale, stopper la transposition des directives européennes. J'insiste sur la nécessité de soumettre les produits importés aux mêmes contraintes que les produits français. Exiger une réelle réciprocité des normes de production témoigne du bon sens. Le texte initial était une forte déception. Le Sénat est mobilisé pour répondre aux grandes attentes des agriculteurs. Souhaitons que le débat soit

je le rappelle, l'agriculture, c'est la nourriture des hommes. Elle concerne aussi l'aménagement du territoire. Je suis élu d'un département rural où l'activité agricole assure la vie

à nos concitoyens, aux consommateurs et inverser la tendance des dernières décennies qui porte toujours plus atteinte à la santé publique. Je pense vraiment que ce texte

ou par accord interprofessionnel- c'est le cas du secteur du lait de vache -, je comprends l'intention et l'importance d'une contrainte forte qui exclut tout contournement de l'accord-cadre par l'acheteur. En revanche, dans les secteurs où la contractualisation écrite n'est pas obligatoire et pour lesquels tant les plans de filières que le projet de loi font mention d'une ambition de développer la contractualisation,

Que le ministre veuille revenir à la rédaction initiale du texte, à rebours du choix de la majorité de l'Assemblée nationale, me semble une bonne chose, car cela donne un peu de souplesse. C'est la raison pour laquelle,

ou de mesures à la marge. Cela fait de trop nombreuses années que des projets ou propositions de loi sont débattus et adoptés sans que rien ne change ! Il n'est qu'à se rappeler les interventions précédentes. Il est nécessaire de remettre en cause la domination sans partage sur la valeur ajoutée au sein des filières de la grande distribution. Il faut mettre un terme à la déréglementation des relations commerciales et remettre en cause le principe même de libre négociation des conditions générales de vente qui a affaibli les producteurs dans les négociations. Lors des États généraux de l'agriculture, ce constat a été unanimement reconnu : si l'on veut sauver l'agriculture française, l'amener vers plus de qualitatif, il faut des prix minimaux garantis. On a besoin dans ce pays de régulation, et cela fait environ trente ans que l'agriculture est la variable d'ajustement à la guerre des prix.

planchers d'achat aux producteurs pour chaque production agricole, en tenant notamment compte de l'évolution des coûts de production, du système de production et des revenus agricoles sur chaque bassin de production.

pour permettre un rééquilibrage des relations commerciales dans le monde agricole. Cela permettra, par exemple, de contrer la grande distribution, qui organise une politique active d'importation et de promotion en fonction de l'arrivée des productions françaises sur les marchés, pour faire pression à la baisse

lequel nous indique : « les prix payés aux agriculteurs ont été à nouveau inférieurs à la réalité des coûts de production et n'ont pas couvert la rémunération du travail ni du capital, et cela même en tenant compte des aides européennes ».

permettant de rééquilibrer les relations commerciales entre producteurs agricoles et acheteurs. Si nous n'aboutissons pas à un accord sur ce sujet, alors la future loi pourra être considérée comme un simple « enfumage

précédents, vise à revenir sur l'un des fondamentaux des États généraux de l'alimentation : garantir un revenu à nos agriculteurs. Dans son discours de Rungis, le Président de la République s'était engagé à modifier

indicateur relatif aux coûts de production, l'objectif d'une juste rémunération du producteur assurée par le dispositif de la contractualisation ne pourra en aucun cas être atteint. Je veux

Reprenant une proposition de la Confédération paysanne, et en cohérence avec nos amendements précédents, nous souhaitons simplifier et réformer. Vous voyez, monsieur le ministre, que nous aussi, nous sommes en marche, ... Bravo ! ... mais vers le progrès social

ces indicateurs et comment les rendre publics, afin que les opérateurs puissent s'y référer ? Nous ne nions pas les améliorations rédactionnelles apportées par la commission des affaires économiques du Sénat et le renforcement du rôle consultatif de l'Observatoire

indépendante des différents acteurs. Il est primordial qu'ils soient déterminés par un organisme public et qu'ils soient acceptés par toutes et tous. et tous. Ils doivent s'appuyer sur des chiffres provenant, notamment, des interprofessions et des instituts techniques agricoles, mais il reviendra à l'Observatoire de proposer les indicateurs de référence servant à la construction si l'on fait reposer les prix de vente sur une multitude d'indicateurs mesurant des choses différentes, ceux-ci finiraient par s'annuler entre eux, chacun utilisant celui qui va dans son intérêt ou le construisant lui-même. Cela ne permettrait pas une juste rémunération des productrices et producteurs.

Cela passe par la construction du prix de vente à partir des coûts de production. Or dans la version actuelle du projet de loi, il est prévu que ce prix de vente prenne en compte aussi bien des indicateurs de coûts de production du paysan français que les prix de vente sur des marchés où opère l'acheteur,

prix. Laisser aux interprofessions l'élaboration et la diffusion d'indicateurs adaptés à leur filière est une avancée, mais nous proposons d'aller plus loin pour sécuriser et rendre plus neutres et indiscutables les prix, tout comme ces indicateurs. Le présent amendement vise donc à rappeler le caractère public des indicateurs et à en confier la définition à l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. L'Observatoire a pour mission d'éclairer les pouvoirs publics sur la formation des prix. Il étudie les coûts de production, les coûts de transformation, les coûts de distribution et examine la répartition de la valeur ajoutée tout au long de la chaîne de commercialisation des produits agricoles. Il a donc toute compétence, mais aussi la légitimité pour produire les meilleurs indicateurs publics. Très

Pendant les États généraux de l'alimentation, nous avons mis en avant la nécessité de responsabiliser les interprofessions. C'est un objectif important. Il est tout aussi important que les OP puissent conserver la possibilité de proposer à leurs acheteurs des indicateurs adaptés à leur situation, en tenant compte des caractéristiques de leur production, ainsi que de la stratégie qu'elles veulent poursuivre. Si l'on considère la filière laitière, par exemple, le coût de production et de

messieurs les sénateurs, à inverser la contractualisation et à rééquilibrer le rapport de force au sein de la filière. Pour cette raison, nous avons soutenu plusieurs amendements concernant les articles 4 et 5 , nous y reviendrons plus tard. Ces dispositifs contribueront à éviter qu'une partie

mais en empruntant un chemin différent, c'est-à-dire en faisant en sorte que les OP soient prééminentes. Ainsi, afin de garantir la liberté contractuelle, la négociation libre et volontaire par les OP, mais aussi de placer les OP et les AOP en responsabilité, il convient de s'assurer que le choix des indicateurs reste le plus ouvert possible au sein d'un panel d'indicateurs disponibles, et ce au bénéfice des producteurs, qui peuvent en être eux-mêmes auteurs. S'il faut saluer la mise en place de ces indicateurs, et surtout la construction du prix autour d'eux, ces indicateurs ne doivent pas, d'après moi, devenir des carcans ou revêtir une dimension contraignante pour les producteurs. Il paraît dès lors nécessaire de réinscrire dans le texte du Sénat la rédaction positive issue des travaux de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale qui prévoyait que « les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles. » Les indicateurs conservent ainsi leur vocation à éclairer les parties dans leur choix, ce qui ne peut que contribuer à renforcer le rôle des OP dans leur expertise et à améliorer l'équilibre de la relation contractuelle. À cet égard, je pourrais reprendre votre argument concernant l'OP ou les AOP de la filière laitière.

reçoivent un avis de l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires. Il ne s'agit pas de remettre en cause la logique actuelle du texte qui consiste à donner un rôle moteur aux organisations interprofessionnelles, en leur laissant l'initiative de la proposition de ces indicateurs. Nous sommes favorables à cette démarche, nous l'avons déjà dit, qui leur donnera davantage de pouvoirs, mais aussi de responsabilités. Toutefois, nous pensons que certaines organisations interprofessionnelles seront moins bien armées que d'autres pour définir leurs indicateurs et les défendre, le cas échéant. C'est la raison pour laquelle il nous semble intéressant que l'Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires émette des avis, non contraignants, sur la pertinence de ces indicateurs, notamment au regard de l'objectif d'une juste rémunération des producteurs. Ces avis permettront, si nécessaire, de renforcer le choix des interprofessions, en leur donnant une forme de caution de la part d'un organisme public. Nous avons bien conscience, comme nous l'a rappelé le rapporteur en commission,

à éviter qu'un acheteur en position de force n'impose un indicateur, ce qui entraînerait de fait un déséquilibre dans la fixation d'un prix juste payé aux producteurs. La notion d'équilibre entre les parties est, à nos yeux, très importante, car elle est la condition qui permettra au dispositif de contractualisation de fonctionner correctement, c'est-à-dire sans léser les producteurs.

Le projet de loi a, certes, été amélioré en permettant que l'Observatoire propose ou valide un indicateur, en cas d'absence d'accord professionnel. Mais il y a un fort besoin de renforcement du contrôle de cet acteur pour encourager le recours aux indicateurs équilibrés. Rappelons que, au sein des interprofessions, l'aval conserve un droit de veto. Cet amendement a donc pour objet d'éviter que l'acheteur en position de force n'impose un indicateur, source de déséquilibre dans la fixation d'un prix juste payé au producteur.

Ce n'est pas impossible ! Il le retirera ! Certaines OP pourront utiliser leurs propres indicateurs s'ils sont validés par l'Observatoire. J'ajoute que la liberté contractuelle

élaborer ». Cela sous-entend que les industriels et la grande distribution pourraient, eux-mêmes, proposer des indicateurs établis par leurs propres experts. Nous ne

se coordonner et se mettre d'accord pour parvenir à une plus juste répartition de la valeur ajoutée. Donc, il est de notre rôle de leur donner tous les outils pour tendre vers ce but, pour les inciter à faire converger leurs intérêts. Pour autant, pensez-vous qu'il est de notre rôle, du rôle de l'État, de se substituer à ces négociations ? Pensez-vous qu'un organisme pourra prendre en compte à lui seul toutes les spécificités des coûts de production d'une filière ? Pensez-vous que ce même organisme permettra la mise en place de contrats efficients sans désavantager une partie du contrat ?

La nouvelle rédaction de l'article 1 proposée par le Gouvernement respecterait cette vision selon laquelle les filières prennent leurs responsabilités.

d'écrire à la place : « Les organisations interprofessionnelles diffusent les indicateurs choisis qui peuvent être ceux construits par les organisations de producteurs ou les associations de producteurs elles-mêmes.

l'amendement n° 45. Par cet amendement, nous proposons de briser un des obstacles à la transformation de la production agricole française en introduisant une clause permettant de ne pas appliquer d'indemnité de résiliation de contrat en cas de passage à un mode de production biologique. En effet, le monde agricole change ; de plus en plus, les agriculteurs se tournent vers des modes de production responsables, respectueux des sols, de l'environnement, de la biodiversité et des citoyens. Il nous semble donc essentiel d'accompagner cette transformation de la production voulue par nombre de producteurs et de consommateurs en levant le maximum de freins possible, transformation utile également pour l'amélioration du revenu paysan. La production biologique est déjà trop peu soutenue en France ; retirer les entraves à la liberté de choisir le type de production nous semble un minimum pour assurer l'indispensable transition agricole. La

cet amendement, nous proposons de ne pas appliquer d'indemnité de résiliation de contrat en cas de modification du mode de production vers une production biologique. Vous l'avez compris, mes chers collègues, nous souhaitons encourager la transition vers des modes de production biologique en ne pénalisant pas les agriculteurs qui décident de s'engager dans cette voie.

de contrat ou d'accord-cadre écrit comporte une clause permettant de ne pas appliquer l'indemnité de résiliation dans le cas de la conversion d'une exploitation vers le bio. L'amendement n° 490 rectifié, présenté

Or le bio constitue parfois une porte de sortie pour les producteurs en difficulté, qui vont vers ce mode de production pour retrouver du revenu. Comment accepter qu'un producteur, dont l'équilibre économique de l'exploitation est parfois fragile, qui va vers un mode de production à la fois bénéfique pour son exploitation, mais aussi pour l'ensemble de la société soit tenu de payer une telle indemnité ? Cette mesure a été rejetée par l'Assemblée nationale, les députés invoquant la liberté contractuelle. Mais je tiens à rappeler que la Cour de justice de l'Union européenne établit que le droit européen n'empêche pas les États membres d'appliquer des règles nationales qui ont un objectif d'intérêt général, même si ces règles sont susceptibles d'avoir une incidence sur le fonctionnement du marché. Peut-on nier que l'agriculture biologique représente l'intérêt général ? La protection de l'environnement est un principe que nul ne conteste et qui est consacré par le traité de l'Union européenne et par notre Constitution. Or l'agriculture biologique protège notre environnement, toutes les études le montrent et le droit européen le reconnaît explicitement. Cette disposition est donc compatible avec la réglementation européenne. On m'a aussi opposé la rupture d'égalité, mais l'agriculture biologique n'est pas n'importe quel système : elle s'appuie sur un cahier des charges européen et est reconnue comme répondant à un droit fondamental, celui de jouir d'un environnement sain. Monsieur le ministre, je ne comprends pas que l'on puisse, d'un côté, programmer des plans de développement de l'agriculture biologique, inscrire des objectifs de surfaces bio dans ce projet de loi, proposer un plan de sortie des pesticides, et, de l'autre, continuer à autoriser des pratiques qui freinent les conversions. Nous devons limiter la liberté contractuelle face à l'intérêt général.

Nous proposons qu'une conversion à l'agriculture biologique ne puisse entraîner d'indemnités de résiliation de contrat dès lors que l'acheteur est informé dans un délai raisonnable de cette conversion. Nous avons fixé ce délai à un an, mais, monsieur le ministre, nous sommes ouverts à la discussion si vous êtes prêt à soutenir cet amendement.

la libre négociation des éléments du contrat, notamment les clauses de résiliation, ce qui interdit aux États membres de priver totalement les parties de la possibilité de prévoir de telles indemnités dans leur droit national. Même si je

Monsieur Labbé, mesdames, messieurs les sénateurs qui avez défendu ces amendements, je partage totalement cet objectif de défense et de promotion de l'agriculture biologique. D'ailleurs, j'ai donné un avis favorable sur un amendement des députés qui visait à ce que le délai de préavis et l'indemnité préalable applicable soient réduits en cas de modification du mode de production. Cela figure dans le projet de loi. Mais imposer

la relation contractuelle pour déterminer à la fois le meilleur prix, le meilleur cahier des charges pour la meilleure qualité possible et pour faire en sorte que le prix qui sera fixé entre un acheteur

balance commerciale. Cette agriculture conventionnelle, nous devons la défendre, nous devons travailler sur la recherche, nous devons vendre du boeuf en Chine et ailleurs, parce que c'est cela qui produit de la valeur ajoutée et qui donne de la rentabilité à nos exploitations.

explication de vote. Nous venons d'avoir une discussion sur les meilleurs moyens de rééquilibrer le contrat en faveur du producteur,

mais il me semble important de ne pas avoir une approche idéologique de ces problèmes. Si nous voulons faire comprendre aux transformateurs qu'il est nécessaire que le prix de revient moyen soit pris en compte sur des bases objectives, ne chargeons pas la barque en rendant plus difficile l'exécution des contrats.

Les étapes de négociation entre fournisseurs et distributeurs dominent les filières agroalimentaires et le pouvoir de marché n'est pas équilibré (au détriment des agriculteurs et des consommateurs, qui subissent les baisses de prix pour les premiers et les hausses de prix pour les seconds). Dix ans après, ce constat est toujours d'actualité, preuve que la production agricole ne peut être soumise aux seules lois du marché et qu'il est urgent de remettre en place des mécanismes pour lutter contre l'opacité en matière de fixation des prix agricoles. L'une des préconisations du rapport précité était d'ailleurs d'assurer une plus grande transparence dans la formation des prix au stade de la production, de la transformation et du commerce, ce qui implique une identification claire des marges de chacun des acteurs. Tel est le sens de notre amendement, qui vise à garantir que, lorsque les contrats sont conclus, les prix déterminés ou déterminables reposent sur des critères clairs, lisibles et rendus publics, afin que les exploitants aient une parfaite connaissance des modalités de calcul. Vous le savez, les acheteurs sont des spécialistes de la règle à calcul, et se moquent bien des conséquences concrètes que peuvent avoir leurs règles dans la vie de nos exploitations.

Malgré la sacro-sainte liberté contractuelle, monsieur le ministre, il ne nous semble pas normal qu'un producteur ne parvienne pas à comprendre comment le prix a été déterminé. Il est essentiel que les pouvoirs publics aient une connaissance des prix fixés dans la proposition de contrat ou dans l'accord-cadre, afin de garantir à la fois l'équilibre et la transparence, dans le cadre de la relation commerciale entre un producteur et un acheteur. La parole

Il n'est pas normal qu'un producteur n'arrive pas à comprendre comment le prix a été déterminé. Avec une formule claire, précise et accessible, les instances publiques ayant connaissance du contrat peuvent facilement suivre l'évolution des prix, sur la base de l'évolution des indicateurs utilisés. Il s'agit, selon nous, d'une question d'honnêteté. Quand j'étais professeur et que je donnais des contrôles à mes élèves, je leur communiquais le barème. Cela me paraissait relever de la moindre des honnêtetés et de la pédagogie la plus élémentaire. Quel est

notamment quant à la négociation de clauses de partage de valeur par les agriculteurs ou par leurs associations. Cette disposition est une avancée importante pour le pouvoir de négociation des agriculteurs. Toutefois, il ne faut pas confondre clause de renégociation et clause de répartition de la valeur, dont les objectifs ne sont pas tout à fait similaires.

AOP représentant 2 600 producteurs, 1,2 milliard de litres de lait et 40 % des besoins de Savencia.

a permis d'intégrer des dispositions positives à ce sujet, issues du règlement européen, notamment, la mise en place de clauses de partage de valeur par les agriculteurs ou par leurs associations.

aux clauses tant de renégociation que de répartition de la valeur, dont les objectifs ne sont pas tout à fait similaires. Sans revenir sur la nécessité de prévoir dans les accords-cadres des clauses de renégociation des contrats,

Gontard. De manière assez logique et pragmatique, nous proposons de restreindre aux normes réglementaires en vigueur les obligations de calibrage contenues dans le cahier des charges des professionnels de l'alimentation. de l'alimentation. Instauré dans les règlements européens pour faciliter les échanges commerciaux, le calibrage a été réduit en 2009, pour se limiter à dix types de fruits et légumes. Pourtant, ces normes sont toujours incluses de manière abusive dans de nombreux cahiers des charges, notamment dans la grande distribution. Il en résulte un gaspillage titanesque de produits alimentaires, qui sont directement jetés aux ordures. Selon une étude de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture datant de 2011, le gaspillage alimentaire européen, pour la seule production, est supérieur à 160 kilogrammes par personne et par an. Il est inimaginable qu'un tel gaspillage soit autorisé quand des millions d'êtres humains sont mal nourris, que les agriculteurs peinent à vivre et que les ressources agricoles sont de plus en plus limitées ! Il est temps de sortir de cet artifice de la société de consommation où les légumes et les fruits sont normés et sans défaut. La notion de perfection n'existe pas en agriculture, pas plus que dans le reste du vivant. D'ailleurs, la forme parfaite d'un fruit, si elle fait joli sur un étal, ne garantit en rien sa qualité. La nature n'est pas uniforme ; ainsi, une tomate peut être déformée. Bien plus, la diversité des formes est gage de qualité. Il faut redonner, en quelque sorte, la vérité des aliments à nos concitoyens Enfin, les agriculteurs seront les premiers bénéficiaires de cette mesure, puisque la fin du calibrage leur permettra de vendre plus en gaspillant moins.

de différenciation et de montée en gamme que nous appelons de nos voeux. Par ailleurs, les contrats visés ne peuvent pas avoir d'incidence dans la lutte contre le gaspillage alimentaire. Enfin, supprimer le calibre dans les contrats et laisser les distributeurs

l'inversion de la relation contractuelle et la construction du prix, afin de mesurer concrètement ses conséquences en termes de répartition de la valeur ajoutée entre les producteurs et les industriels. Nous avons bien conscience qu'il appartient au Parlement de suivre l'application de la loi, mais nous connaissons également les difficultés que nous rencontrons pour mener à bien cette mission d'évaluation et de contrôle, tant son étendue est importante. Réformé par ce projet de loi, l'Observatoire

la mission d'évaluation des politiques publiques doit être assumée pleinement par le Parlement, avec ses moyens. Reste que le Parlement ne pourra pas l'exercer de manière complètement autonome, sans travailler avec des organismes extérieurs. S'agissant du sujet qui nous intéresse, c'est bien l'Observatoire de la formation des prix et des marges

Face aux risques d'insécurité juridique, il convient de supprimer la prérogative de définition de ces modalités par les interprofessions. Quel

Le plan de filière de la viande bovine française, réalisé par Interbev à la demande du Président de la République, fixe un objectif ambitieux en matière de développement de la production et de la commercialisation des viandes bovines sous signe d'identification de la qualité et de l'origine, la filière s'est engagée à commercialiser 40 % de viandes bovines sous label rouge d'ici à cinq ans. Cette montée en gamme ne sera possible qu'à travers un encadrement strict des relations commerciales au sein de la chaîne d'approvisionnement de ces viandes sous SIQO, incitant les producteurs à s'engager dans cette voie. C'est pourquoi, alors que la filière viande bovine française n'est pas soumise à contractualisation obligatoire, les auteurs de cet amendement proposent d'encourager l'interprofession à rendre obligatoire à très court terme la conclusion de contrats de vente et accords-cadres écrits mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime spécifiquement pour les viandes bovines commercialisées ne proposons nullement d'imposer cette évolution aux interprofessions, qui travaillent aujourd'hui librement, mais avec des difficultés liées à leur mode de fonctionnement, à la bonne application de leur plan de filière. Quel est l'avis de la commission ?

est à M. Cyril Pellevat. La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, dite loi Sapin II, a créé un dispositif devant permettre une meilleure transparence pour les acteurs du secteur concernés par la contractualisation obligatoire. obligatoire. Pour des raisons de calendrier, elle s'est effectivement appliquée pour les négociations commerciales de 2018 entre transformateurs et acheteurs. Le présent projet de loi intervient moins d'un an après l'entrée en vigueur effective de la loi Sapin II. de la loi Sapin II. S'appuyant sur les conclusions des États généraux de l'alimentation, il doit compléter et renforcer les dispositions de la loi précitée. Il est donc proposé de laisser vivre le dispositif instauré pour la contractualisation rendue obligatoire, mais également de créer une sanction dans le cas où le prix prévisionnel moyen n'est pas indiqué dans les conditions générales de vente. Nous

Monsieur le ministre, vous avez dit que les

proposition du dispositif de cascade : les indicateurs présents dans les contrats, c'est-à-dire ceux qui sont utilisés dans la détermination du prix du producteur, seront pris en compte dans chacun des contrats passés ensuite avec un acteur en aval de la filière. Il s'agit de tirer les leçons de l'application de la précédente loi, bien qu'elle soit très récente, et de proposer un dispositif d'une plus grande efficacité. Pour cette raison, je suis défavorable à cet amendement.

Or, en cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l'acheteur, la sortie du contrat doit être facilitée, afin de favoriser la montée en gamme de l'agriculture et de ne pas pénaliser les producteurs qui changent de système.

aller encore plus loin en exemptant les coopératives d'indemnités réduites en cas de changement de mode de production est tout simplement injustifié. La montée en gamme de notre agriculture est l'un des moyens de garantir un revenu à nos agriculteurs et la recherche de valeur ajoutée est également bénéfique pour l'environnement, la vie dans nos campagnes, la qualité de l'alimentation. Nous devons donc défendre les producteurs, les territoires, la biodiversité et choisir de lever tous les freins qui empêchent les producteurs d'aller vers des systèmes vertueux. L'amendement

est à M. le ministre. Le texte adopté par la commission des affaires économiques du Sénat exclut pour les coopératives la définition d'une clause relative aux délais de préavis et à l'indemnité applicable lors de la résiliation du contrat. Pourtant, la sortie du contrat coopératif ou le retrait de l'associé coopérateur sont prévus par les statuts coopératifs et ne peuvent qu'exceptionnellement intervenir avant la fin de la période d'engagement du coopérateur. Il ne s'agit pas d'y porter atteinte, mais seulement de prévoir que les délais et les pénalités qui demeurent à l'appréciation du conseil d'administration doivent, en coopérative comme dans le cas général, tenir compte des situations dans lesquelles le départ de l'associé coopérateur est lié

a eu raison de citer les 550 cas de coopératives qui ont accompagné la mutation vers le bio. Quand il y a eu jugement, le tribunal a fait référence

de la solidarité, et pas du rapport commercial

fasse référence aux indicateurs mentionnés dans le pacte coopératif et non aux indicateurs utilisés pour la rémunération des producteurs associés coopérateurs. En effet, la notion de rémunération est

124 rectifié Cet amendement vise à assurer aux producteurs de betteraves et de canne à sucre les mêmes garanties qu'aux autres agriculteurs. Les planteurs, dont la rémunération baisse, sont particulièrement intéressés par l'obligation pour le contrat de faire référence aux indicateurs utilisés pour la rémunération de leurs betteraves, et ce d'autant plus que, d'une part, les discussions avec certains fabricants sur le prix définitif des betteraves 2017-2018 sont très tendues, et que, d'autre part, les engagements pluriannuels pris par d'autres fabricants sur un niveau de rémunération des betteraves ne seront pas respectés au vu de la très forte dégradation des prix du sucre ces derniers mois. Si la filière de la betterave sucrière bénéficie d'une réglementation européenne étoffée, en matière de contrats de vente de betteraves, le droit national s'est toujours appliqué sous réserve des règlements européens. Ainsi, l'exclusion des betteraviers et canniers du bénéfice des nouvelles dispositions relatives aux contrats de vente de produits agricoles, au motif que seul le droit communautaire s'appliquerait, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne- compétente pour interpréter le droit de l'Union européenne, selon l'article 267 du traité -selon laquelle « si l'organisation commune des marchés prévoit des règles générales relatives à la vente et l'achat des betteraves, il en ressort cependant clairement que les accords et contrats visés continuent, sous réserve du respect desdites règles générales, d'être régis par le droit national des contrats sous lequel ils sont conclus ». Il est donc particulièrement important dans le contexte actuel de renforcer la contractualisation au sein de la filière, notamment en renforçant le rôle de l'interprofession, qui pourrait fournir des indicateurs et définir les modalités de partage de la valeur, ce que permet le projet de loi en discussion, dans le strict respect du droit de la concurrence.

les avancées contenues dans le présent projet de loi pourraient venir compléter utilement le futur accord interprofessionnel qui s'appliquera à compter de 2020. Ainsi, l'exclusion dont les betteraviers et les canniers font l'objet dans le présent projet de loi n'est pas une nécessité au regard du droit de l'Union européenne et elle n'est pas cohérente avec les réalités que connaît la filière sucrière française.

Depuis 2016, la réglementation européenne prévoit déjà la possibilité d'établir des clauses de répartition de la valeur régies par l'accord interprofessionnel. C'est d'ailleurs ce secteur qui a servi d'exemple à l'ensemble des autres, puisque nous appelons tous de nos voeux le recours à des clauses L'interprofession a mis en place cette clause. Une commission de répartition de la valeur est installée dans chaque entreprise, composée des représentants des planteurs et, bien sûr, des sucriers. Un prix minimal garanti est fixé, avec une prime de revalorisation en fonction des excédents dégagés pour les producteurs. Modifier le régime contractuel applicable à la filière sucrière reviendrait à remettre à plat l'ensemble des accords que celle-ci a conclus et qui semblent plutôt bien fonctionner, malgré l'existence d'un certain nombre de désaccords. Or la remise en cause des clauses de répartition de la valeur semble entraîner plus de risques que d'opportunités. Je suggère que l'on attende de tirer un bilan de cette expérience de trois ans avant de conclure quoi que ce soit.

de déroger par accord interprofessionnel à la loi. Cet amendement tend donc à supprimer cette possibilité, introduite par la commission des affaires économiques du Sénat aux alinéas 48 et 49. Cela étant, il est vrai que les contrats types qui ont été établis par les accords interprofessionnels sont un outil important pour consolider la contractualisation au sein d'une filière. Ils peuvent, par exemple, établir une liste de clauses obligatoires complémentaires ou additionnelles à celles que prévoit le socle de base défini par l'article 1 du projet de loi. Ils peuvent également préciser la rédaction ou le contenu d'une clause type prévue par la loi. Pour répondre à certaines attentes exprimées par les différentes interprofessions, dont celle du secteur vitivinicole, il est proposé de rappeler explicitement cette possibilité dans le texte de la loi, en y indiquant que les interprofessions peuvent préciser et compléter, par accord interprofessionnel, les clauses prévues par la loi. J'ai pu constater, dans les récents échanges que j'ai eus avec certaines interprofessions, que cet ajout était de nature à les rassurer et répondait à leurs attentes. J'ai cru comprendre que leurs représentants vous avaient alertés en nombre,

Il est donc essentiel d'élargir la disposition qui a été adoptée par la commission des affaires économiques au plus grand nombre. Cela permettra à la loi de prévoir le cas d'accords interprofessionnels étendus, tout en répondant à l'objectif initial, à savoir développer la contractualisation.

Afin de prendre en considération ces spécificités, à savoir le caractère météo-sensible, la très grande diversité des produits, la diversité des modes et des coûts de production ainsi que des schémas de commercialisation, il est proposé de laisser à l'interprofession, à partir du moment où elle représente l'ensemble des maillons de la filière, de la production jusqu'à la distribution, la possibilité de préciser, voire de compléter, par accord interprofessionnel, les dispositions de la loi et de prévoir les modalités spécifiques de contractualisation. Cet accord interprofessionnel permettra d'encadrer de manière volontaire la contractualisation, afin de la rendre attractive et adaptée à la filière.

nous avons auditionnées demandaient une telle exonération ! La raison en est probablement que les éléments minimaux à prévoir dans les contrats sont assez souples et acceptables par tous. Un contrat est fait pour protéger un producteur dans sa relation avec l'aval, qui est concentré. Pour ce faire, il convient de prévoir des clauses minimales dans un contrat. Si l'on nivelle par le bas, par le recours aux accords interprofessionnels moins-disants, le risque est d'avoir un effet contre-productif. Il faut donc limiter les dérogations.

Le formalisme est mal adapté à la filière viticole, pour laquelle la plupart des contrats, au demeurant ponctuels, pour l'essentiel, des contrats spot, sont réalisés par l'intermédiaire d'un courtier qui est mandaté par les deux parties au contrat. Or le courtage n'est même pas envisagé dans le projet de loi. Je maintiens donc la position initiale de la commission, et j'émets un avis défavorable sur les trois amendements.

plus particulièrement ceux des distributeurs, sur l'ensemble de la filière. Il s'agit d'une régulation par l'État des prix et du marché. Ce dispositif est déjà l'objet de l'article L. 611-4-2 du code rural et de la pêche maritime, mais il ne concerne actuellement que les fruits et légumes, avec un déclenchement laissé à la libre appréciation des ministres chargés de l'économie et de l'agriculture. Si, depuis l'instauration de ce dispositif, son activation a été évoquée à plusieurs reprises, jamais cette démarche n'a été concrétisée. L'argument de la complexité de ce mécanisme est difficile à entendre, étant donné qu'il existe depuis maintenant des années.

bien évidemment aux périodes de crise conjoncturelle ou en prévision de celles-ci. En s'appliquant également aux produits agricoles importés, cette extension du coefficient multiplicateur constituerait aussi un puissant levier de dissuasion envers les pratiques de mise en concurrence des productions, notamment en fonction de la date d'arrivée sur le marché, et de dumping économique, social et environnemental Nous pensons que ce mécanisme risque de tendre le dialogue entre les acteurs des filières, raison pour laquelle le dispositif de l'amendement précise également que les ministres chargés de l'économie et de l'agriculture devront, avant de décider du taux et de la durée du coefficient multiplicateur, consulter non seulement les organisations professionnelles concernées, mais également les syndicats agricoles. Enfin, la limitation à trois mois de l'application du coefficient multiplicateur est supprimée par le biais de cet

des pratiques abusives des intermédiaires, particulièrement en matière de marges. Nous débattons à son sujet de façon récurrente. L'objectif est bien de permettre la satisfaction des besoins des Français par une maîtrise publique et d'empêcher les spéculateurs de déstabiliser les prix.

Cet amendement vise à lutter contre le chantage à la collecte et le déréférencement des producteurs. En effet, ces deux instruments pervers donnent une force colossale de négociation aux acheteurs industriels. L'inversion de la construction des prix comporte des risques pour les producteurs et cet amendement tend à les protéger de pratiques de négociation abusives et critiquables. La peur de ne plus être collecté place les producteurs dans une position de faiblesse à l'égard de leurs acheteurs, à cause de leur dépendance économique. Conformément aux remarques exprimées par M. le rapporteur en commission et à la suite des échanges avec l'administration, la nouvelle rédaction de cet amendement propose une solution « 3+3 », selon laquelle, outre le délai de préavis à la rupture d'un contrat de trois mois, le producteur de lait ou de denrées périssables dispose de trois mois supplémentaires pour pouvoir, en quelque sorte, se retourner.

pour la bonne et simple raison que, tant que le litige n'est pas réglé, le transformateur doit continuer à collecter, quelle que soit l'issue des négociations.

pour prolonger de trois mois le contrat arrivé à expiration, ce qui est contraire à la liberté contractuelle, j'invite les participants à anticiper les dates de fin de contrat et à commencer la médiation au moins trois mois avant la date d'expiration, maintenant que les délais en la matière sont très encadrés,

L'un de nos objectifs est de permettre aux producteurs de vendre à un prix rémunérateur et de sortir de la précarité des milliers d'agriculteurs. Or, si ce projet de loi vise à une répartition plus juste de la valeur ajoutée, l'un des moyens d'y parvenir est d'informer et de responsabiliser les consommateurs. En effet, en indiquant sur l'étiquette des produits la manière dont est répartie la valeur ajoutée, nous permettons aux Français d'être plus avisés dans leurs achats. Par ailleurs, les consommateurs pâtissent aussi de cette mauvaise distribution de la valeur ajoutée, puisqu'ils sont floués par le prix. Il est fréquent que les prix soient trop élevés et rémunèrent trop le distributeur, ou, à l'inverse, qu'ils soient trop bas et ne rémunèrent pas assez le producteur. Par cet amendement, nous permettons aux citoyens de remédier à cette situation. En effet, consommer est devenu un acte citoyen les Français sont de plus en plus nombreux à adopter un comportement d'achat qui vise à promouvoir des productions locales et responsables, mais aussi les produits dont la valeur ajoutée est équitablement partagée. La croissance constante de la consommation des produits locaux, bio, de saison ou issus du commerce équitable en témoigne.

L'article 2, que nous nous apprêtons à étudier, est d'une importance centrale, puisqu'il permet de sanctionner les manquements aux obligations contractuelles, par la prévention des situations où l'acheteur aurait la tentation de se placer en position de force vis-à-vis d'un ou de plusieurs producteurs. producteurs. Dans ce cadre, nous avons déposé plusieurs amendements, qui visent à redonner de la force à notre législation et, surtout, à faire en sorte que les dispositions coercitives dissuadent de toute infraction tout abus de pouvoir. Dans notre volonté d'une discussion constructive, nous proposerons des mesures échelonnées. D'ailleurs, l'un de nos amendements tend à fixer la sanction à 5 % du chiffre d'affaires. chers collègues, nous devons travailler à une loi qui protège, afin de donner aux autorités compétentes les moyens de défendre les plus faibles face aux plus forts. Nous pensons que, pour que ce texte soit crédible dans sa tentative de permettre aux producteurs de percevoir un juste niveau de rémunération, les amendements

à nos agriculteurs, en leur montrant que nous voulons une contractualisation équilibrée, permettant l'émergence de prix justes et, surtout, l'octroi d'un revenu décent. Nous ne pouvons laisser mourir de faim des femmes et des hommes qui nourrissent les femmes et les hommes de notre pays. Il appartient dès aujourd'hui à la puissance publique de permettre une régulation visant à s'assurer de ce bon équilibre de la relation entre les producteurs et les acheteurs.

442-6 du code de commerce sur les pratiques restrictives de concurrence. Nous voulons rappeler qu'une action peut être introduite devant une juridiction civile ou commerciale compétente, par le ministère public, par le ministre chargé de l'économie ou par le président de l'Autorité de la concurrence lorsque ce dernier constate une pratique restrictive de concurrence. Si une situation illicite est avérée, les autorités compétentes que je viens de citer peuvent faire constater la nullité des clauses ou des contrats illicites et demander la répétition de l'indu.

Et malheureusement, ce texte, qui s'inscrit dans la même logique, n'échappera sûrement pas à cette règle. C'est la raison pour laquelle nous proposons de porter à 5 % du chiffre d'affaires le taux des sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions prévues à l'article 1 du projet de loi, tout en ayant conscience que ces mêmes sanctions pourront désormais s'appliquer aux producteurs. Toutefois, comme l'a souligné le rapporteur, deux adaptations protègent ces derniers : d'une part, contrairement à l'acheteur, le producteur ne sera pas sanctionné s'il propose un contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 d'autre part, les sanctions seront adaptées à la taille des organismes concernés et les petits producteurs n'auront pas à payer les mêmes montants que des acteurs réalisant un chiffre d'affaires de plusieurs milliards d'euros.

tel que modifié par la loi Macron, prévoit des sanctions pouvant aller jusqu'à 5 % du chiffre d'affaires en cas d'atteinte au droit de la concurrence, par exemple, mais aussi en cas de déséquilibre significatif ou de rupture brutale

qui ne leur appartient plus, et cela durant des mois. Mais il y a plus important : certains négociants jouent sur l'importance de ces stocks, à la veille des vendanges, par exemple, pour tenter de renégocier les prix à la baisse sous différents prétextes et même parfois, me précise-t-on, pour remettre en cause les contrats. En l'espèce, c'est donc le pot de terre contre le pot de fer. D'où mon interrogation : que valent, dans certains cas et dans certaines situations, les accords interprofessionnels Face à cette situation, j'avais fait adopter, en 2008, un amendement visant à obliger l'acheteur à verser un acompte de 15 % à la signature du contrat.

Mais les accords interprofessionnels prévoient que des acomptes seront versés tout au long du contrat. En Champagne, par exemple, le prix est réglé en quatre échéances à partir du mois de décembre qui suit la récolte- la dernière intervenant avant la récolte suivante et la première est au moins de 25 %. Dans le Val de Loire, les vins achetés hors contrats pluriannuels sont payés dans les délais de droit commun, l'acompte n'est donc pas une préoccupation essentielle. que les accords interprofessionnels nécessitent l'unanimité et donc l'accord des producteurs. Cela doit faire l'objet de négociations pour que ce délai de versement soit le plus adapté aux contraintes géographiques vinicoles. Pour ces raisons,

Les agriculteurs ne travaillent pas pour rien. C'est la raison pour laquelle nous proposons de sanctionner l'achat de produits en dessous de leur coût de production, déterminé par les indicateurs fournis par l'Observatoire de la formation des prix et des marges. Quel est l'avis de la

l'avis du Gouvernement ?

uniquement à la charge de l'une des parties. Vous l'aurez compris, cela crée une situation de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, alors que rien ne justifie une telle unilatéralité

outre, ce déséquilibre peut constituer une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce. Cet amendement vise donc à sanctionner les pratiques constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs sur la même base que le sont les relations industrie-commerce. La parole est à M. Claude

une pratique restrictive de concurrence sanctionnée par l'article L. 442-6 du code de commerce. Cet amendement vise donc à instaurer une mesure qui relève de la justice à l'égard de nos producteurs, sur l'ensemble de nos territoires. Les pratiques abusives de ce type, constatées entre les producteurs et leurs premiers acheteurs, devront être sanctionnées sur la même base que le sont les relations industrie-commerce.

producteurs de lait. Cet exemple n'est pas anodin, monsieur le ministre. Cet amendement fait d'une pierre deux coups, puisqu'il traite d'une problématique qui concerne aussi bien les relations entre le producteur et son premier acheteur que les contrats en aval.

Ce manquement est difficilement contrôlable par les agents chargés de constater les manquements, puisqu'il comporte une part subjective.

et distributeurs. De plus, les sanctions ne pouvant s'appliquer que lorsque le contrat est en cours, l'acheteur ne peut arrêter la collecte du produit pendant l'exécution du contrat, sous peine de s'exposer à des sanctions. Enfin, en cours de contrat, si le chantage a lieu au moment de la renégociation, le producteur peut invoquer les dispositions de l'article L. 442-6 du code de commerce qui sanctionne le fait de tenter d'obtenir, sous la menace d'une rupture brutale totale ou partielle des relations commerciales, des conditions abusives concernant les prix.

que les conditions de transparence sur le marché facilitent un juste retour au producteur agricole. Il s'agit donc d'organiser une veille de la fonctionnalité du marché agricole et de pouvoir alerter sur un éventuel dysfonctionnement.

qui précise que le médiateur peut, sur demande des ministres de l'agriculture et de l'économie, émettre des recommandations sur les modalités de partage équitable de la valeur ajoutée. La commission demande donc le retrait

Or l'atelier 7 des États généraux de l'alimentation avait conclu à la nécessité de mettre en place un arbitrage public. Il a donc été introduit à l'Assemblée nationale un alinéa permettant au médiateur de saisir le ministre de l'économie en cas d'échec des négociations. Concrètement, cela ne fera qu'ajouter un intermédiaire. Il serait plus judicieux que le médiateur puisse directement saisir le juge quand il l'estime nécessaire. C'est pourquoi, par cet amendement, il est proposé que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse recourir au juge en cas d'échec de la médiation, à condition qu'il justifie de son intérêt à agir. L'amendement

pour faire constater la nullité d'un contrat, non plus lorsqu'il est jugé illicite, comme le prévoit l'amendement du Gouvernement, mais dès que le médiateur a estimé qu'un déséquilibre contractuel persistait. En effet, face au caractère périssable des produits concernés par les contrats, il est impératif, conformément aux conclusions de l'atelier 7 des États généraux de l'alimentation, que la procédure en cas d'échec de la médiation prenne

sens. Le présent amendement tend donc à renforcer l'effectivité de la mesure, en supprimant son caractère facultatif. Dès lors que le médiateur a estimé qu'un déséquilibre contractuel persistait, Enfin, le médiateur des relations commerciales agricoles ayant une double tutelle, il est normal que le ministre de l'agriculture puisse également saisir le juge.

Mais une telle disposition ne va pas assez loin. Il faut également que le médiateur puisse saisir le juge en la forme des référés. En effet, au vu du rapport de force déséquilibré au sein des filières, la possibilité pour un acteur extérieur de saisir le juge est essentielle. Il est nécessaire que le médiateur puisse avoir cette possibilité, pour garantir un recours efficace en cas d'échec de la médiation. Sans possibilité d'arbitrage en cas d'échec de la médiation, le projet de loi restera largement inefficace au regard de l'objectif de répartition équitable de la valeur dans la chaîne alimentaire.

défavorable à l'idée d'obliger le médiateur à saisir le ministre s'il constate une clause instaurant un déséquilibre manifeste. Le rôle premier du médiateur dans un litige est de trouver une conciliation entre les parties. S'il doit automatiquement transférer tous les litiges au niveau du ministre, ce n'est plus de la médiation, mais un contrôle administratif. En outre, cela contribuera à empiler les parapheurs sur le bureau du ministre, au détriment de son sommeil

préjudiciable à la qualité des relations commerciales et à la mission du médiateur. Toutefois, compte tenu d'un rapport de force déséquilibré dans certains cas, je partage l'objectif recherché, à savoir

la possibilité pour le médiateur de saisir le ministre chargé de l'économie de toute pratique qu'il estime présenter un caractère abusif, afin que celui-ci puisse, si nécessaire,

puisse alerter d'un déséquilibre dans le dispositif de contractualisation. Quel

En effet, ces derniers s'autorisent trop souvent à mettre fin à la collecte des produits lorsque les négociations sur le contrat échouent. Dans le cas de produits rapidement périssables comme le lait, cela a pour conséquence de mettre sous pression les producteurs, qui craignent de ne plus être collectés et de perdre leur production, ce qui les place en position de faiblesse dans la négociation. Ainsi, afin de sortir des milliers d'agriculteurs de la précarité et de leur permettre de dégager un prix rémunérateur pour leur activité, nous proposons d'interdire la cessation de collecte lors de la négociation des contrats, tout en précisant que le contrat précédent reste en vigueur en cas de blocage dans la négociation.

au-delà de la date d'expiration, ce qui est contraire à la liberté contractuelle, il faut anticiper les dates, ce que nous avons fait tout à l'heure, en adoptant des amendements en ce sens. Le Gouvernement est donc défavorable à ces amendements.

Le plus souvent, le litige concerne l'élaboration de la formule de prix, la révision ou la négociation de ce prix. Le taux de réussite de l'intervention est actuellement de 30 %, ce qui est significatif. Toutefois, un renforcement du rôle et des actions du médiateur pourrait permettre un meilleur taux de règlement.

l'issue d'une médiation peut avoir valeur d'exemple. Cet amendement vise donc à supprimer cet accord des parties, pour rendre le dispositif plus efficient.

souligner une situation de blocage imputable à l'une ou l'autre des parties ou aux deux parties. Cependant, seul le médiateur est en capacité de décider s'il doit publier les éléments, et il n'est pas pertinent de demander l'accord des parties. En effet, si l'une des parties est à l'initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu'elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c'est effectivement dans ces situations que la procédure est utile. L'amendement permet de ne pas enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. L'amendement ainsi libellé : La parole est à M. Fabien Gay. Le médiateur des relations commerciales agricoles peut être saisi en cas de litige relatif à la conclusion ou à l'exécution d'un contrat de vente ou pour donner un avis sur toute question relative aux relations contractuelles entre les acteurs d'une filière. Cet amendement vise donc à permettre que la publication des conclusions d'une médiation ait valeur d'exemple pour l'ensemble des opérateurs placés dans une situation comparable.

Dans ce cas précis, seul le médiateur doit être en capacité de décider s'il doit publier les éléments. Il n'est pas pertinent de demander l'accord des parties. En effet, si l'une des parties est à l'initiative du blocage de la médiation, il est bien évident qu'elle ne permettra pas la publication des conclusions. Or c'est effectivement dans ces situations que la procédure est utile. L'amendement permet de ne pas enfreindre l'obligation de confidentialité attachée à toute médiation par la loi du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative. L'amendement

est ainsi libellé : La parole est à Mme Angèle Préville. Cet article vise à permettre au médiateur des relations commerciales agricoles de rendre publiques ses conclusions en cas de litige. La rédaction actuelle de l'alinéa 11 prévoit que cette publication ne pourra se faire que « sous réserve de l'accord préalable des parties Or il est évident que les parties concernées, à commencer par les auteurs d'éventuelles infractions ou conduites condamnables, refuseront de donner leur accord. En conséquence, maintenir l'accord préalable des parties détourne le dispositif initial de son objectif, à savoir la dissuasion, et le rend inopérant. il s'agit de cibler et de dénoncer les entreprises qui ne jouent pas le jeu et ont des comportements condamnables, le présent amendement s'inscrit dans la logique de ce projet de loi, en donnant une véritable effectivité au . Quel est

ans, 7 médiateurs internes aux enseignes. Ils ont traité 45 dossiers sur 60 litiges entre fournisseurs et distributeurs. Pour soutenir cette capacité de règlement des litiges, cet amendement prévoit que le médiateur des relations commerciales agricoles puisse, le cas échéant, déléguer des litiges au médiateur interne des entreprises,

En outre, une telle autoévaluation, si elle est suivie de propositions d'améliorations, nous semble profitable à l'heure où nous souhaitons améliorer le contrôle et renforcer la bonne application de la loi.

Or il a été répété à l'envi qu'il était nécessaire d'assurer une montée en puissance d'un tiers impartial et indépendant et que l'action du médiateur des relations agricoles serait centrale dans la réussite du dispositif adopté à l'article 1. Les relations économiques au sein des filières agricoles sont déséquilibrées, toujours au bénéfice de l'aval. Les agriculteurs sont en position de faiblesse par rapport à leur premier client. Les transformateurs, eux, le sont par rapport aux distributeurs ou aux grandes chaînes. Compte tenu du rapport de force actuel, il est difficile d'imaginer qu'une autre médiation soit efficiente. Pour reprendre les mots de la plaquette d'information disponible sur le site du médiateur, l'accompagnement par un médiateur formé aux négociations est un gage de réussite pour les parties qui souhaitent trouver un terrain d'entente. Le médiateur n'est ni un juge ni un arbitre ; il s'engage et s'astreint à respecter des principes établis et reconnus : confidentialité, indépendance, impartialité et neutralité. L'amendement n°

qui viennent d'être défendus. Cet amendement prévoit la possibilité de passer par un autre dispositif de médiation, dès qu'il est prévu par le contrat, sans exigence d'une équivalence du dispositif de médiation. Ce point est important, car certaines filières, comme les céréales ou le sucre,

dont nous avons discuté avec la FNSEA, que les recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles soient utilisées par le juge en cas d'échec de la médiation. Ainsi, le juge pourra prendre une décision en la forme des référés se fondant sur les conclusions du médiateur sans pour autant rouvrir tout le dossier. Cela représente un gain de temps considérable, notamment pour la partie qui a

mais il fallait aller plus loin. C'est pourquoi un jugement en la forme des référés, qui n'est pas un référé- un référé se contente de bloquer un litige en l'attente d'un jugement sur le fond -, permettra à un juge de statuer rapidement au fond sur le litige en cas d'échec de la médiation, qui demeure un préalable à toute saisine du juge. Ces délais induisent évidemment que le juge s'appuiera sur l'ensemble des pièces disponibles, un peu comme un juge s'appuie sur les conclusions des avocats. Le juge est souverain dans sa décision. Il doit pouvoir juger sur l'ensemble des pièces qui lui semblent utiles. Les conclusions du médiateur, dont l'indépendance est reconnue, seront évidemment au coeur du dossier, mais ce ne seront pas les seules pièces potentielles si le juge estime qu'il a besoin d'éléments complémentaires.

sur ces amendements. Quel est l'avis du Gouvernement ? Le fait de statuer sur la base de l'avis du médiateur implique une transmission automatique des recommandations du médiateur au juge. Dès lors que cette disposition ne renvoie pas à l'accord des parties, ce point n'est pas compatible avec la confidentialité de la médiation.

L'idée était de créer, comme le prévoyait d'ailleurs une des propositions de l'atelier 7 des États généraux, une commission d'arbitrage qui fonctionnerait comme une juridiction à part entière, sa décision s'imposant à tous les acteurs. Il s'agissait d'instaurer une culture de la négociation qui aboutisse au préalable de cet arbitrage public. Un des arguments avancés pour rejeter ces amendements était que la création de cette nouvelle commission d'arbitrage aurait constitué une nouvelle juridiction étatique spécialisée de l'ordre judiciaire et que cette commission aurait été compétente en lieu et place des juridictions de droit commun pour connaître des litiges persistant à l'issue de la médiation engagée sous l'égide du médiateur des relations commerciales agricoles. Enfin, dans son principe, une telle option s'écartait de l'orientation générale du chantier de simplification de l'organisation judiciaire et de la procédure civile en cours d'étude par le Gouvernement. Cet amendement, que nous avons travaillé avec la Confédération paysanne, vise à confier une mission d'arbitrage à la Commission d'examen des pratiques commerciales ; il n'y a donc pas création d'une nouvelle juridiction. Cela donne au contraire à la médiation une chance d'aboutir. L'objectif est d'avoir un pouvoir dissuasif à terme plus important que le pouvoir d'arbitrage en soi, afin que les relations commerciales agricoles s'apaisent d'elles-mêmes par l'instauration d'une culture de la négociation